L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979,

le 6 décembre 2019, la France et l'Argentine ont signé un avenant à la convention du 4 avril 1979 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, déjà modifiée par un avenant en date du 15 août 2001. Cette convention, qui fut le second instrument signé par la France avec un pays membre du Mercosur, témoigne des relations fluides et solides qu'entretiennent nos deux pays depuis de nombreuses années. années. Elle fixe les règles de répartition du droit d'imposer entre la France et l'Argentine, dans le but d'éliminer les doubles impositions pouvant résulter de l'application des législations fiscales nationales sur les différentes catégories de revenus qu'elle vise.

La conclusion de cet avenant s'inscrit dans le cadre d'une excellente relation bilatérale, qui investit de nombreux domaines : produits pharmaceutiques, parfumerie, chimie organique de base, agriculture, automobile. Ainsi, le dialogue politique entre nos deux pays s'est considérablement développé ces dernières années, comme en témoignent les entretiens réguliers entre les ministres des affaires étrangères et la visite du président Fernandez en France, au mois de février 2020.

que l'avenant à la convention fiscale aujourd'hui proposé à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, permettra encore de développer. Je souhaite maintenant vous présenter les avancées permises par la conclusion de cet avenant. Tout d'abord, conformément à l'objectif visé par la France, cet avenant réduit les taux plafonds conventionnels de retenue à la source sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et les gains résultant de la cession d'actions. Cette réduction se fera au bénéfice du Trésor public français, à la charge duquel le montant de l'impôt argentin à éliminer sera diminué. Compte tenu de l'asymétrie des flux d'investissement, qui se traduisent par une forte présence des entreprises françaises en Argentine, l'abaissement de ces taux joue mécaniquement en faveur de nos intérêts économiques

permet également de lutter contre les schémas d'évasion fiscale lors de la cession d'immeubles au travers de fiducies ou de trusts. Il précise, en outre, le champ d'application des redevances taxables en Argentine,

En échange de ces avancées, la France a accepté l'insertion d'une clause relative aux établissements stables, c'est-à-dire d'une base taxable, en l'absence de toute installation matérielle, dès lors qu'une entreprise rend des services dans un État pour une durée représentant plus de 183 jours au cours d'une année. clause est présente dans la quasi-totalité des conventions signées par l'Argentine, ainsi que dans de nombreuses conventions fiscales conclues par la France.

La présence française en Argentine demeure aujourd'hui significative, puisque 15 000 de nos ressortissants y sont établis, notamment près de 1 000 étudiants. La France figure au huitième rang des investisseurs étrangers en Argentine, tandis que de grands groupes français y sont implantés, ainsi que près de 250 entreprises.

Depuis la signature d'un avenant en 2001, les intérêts, les dividendes et les redevances sont en principe imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Néanmoins, la convention autorise l'État d'où proviennent ces revenus à taxer ces derniers, dans la limite d'un plafond fixé à 15 % pour les dividendes, à 20 % pour les intérêts et à 18 % pour les redevances. Cette retenue à la source ouvre droit, en France, à un crédit d'impôt équivalent, qui ne peut excéder l'impôt dû en France au titre de ces revenus. Les gains en capital, quant à eux, font l'objet d'un traitement différent, puisqu'ils sont exclusivement imposables dans l'État source, sans que cet impôt soit plafonné. À l'aune de ces éléments, notamment des taux élevés de retenue à la source, il apparaît que la convention franco-argentine se rapproche davantage du modèle de convention de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui vise à octroyer aux pays en développement plus de droits d'imposition sur les revenus générés par les investissements étrangers qui y sont réalisés.

en renchérissant le coût des investissements pour les entreprises françaises, d'autre part, en diminuant les recettes fiscales pour le Trésor public. De plus, rien ne justifie le maintien de ces taux, l'Argentine ayant conclu ces dernières années des conventions fiscales nettement plus avantageuses, qui prévoient des plafonds de retenue à la source inférieurs.

Nos négociateurs ont également obtenu l'insertion de plusieurs clauses du modèle France au sein de la convention, ce qui nous permet de continuer à appliquer notre législation interne dans un certain nombre de cas.

Trois avancées significatives ont été obtenues par la France au titre des négociations, à savoir la réduction des taux de retenue à la source, l'insertion de clauses du modèle France et l'élargissement de la clause de la nation la plus favorisée. L'article 2 prévoit une diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15 % à 10 % en cas de participation substantielle du bénéficiaire sur une période de 365 jours.

L'article 3 réduit le taux de retenue à la source sur les intérêts de 20 % à 12 %, soit à un niveau plus conforme au modèle de convention de l'OCDE, qui le fixe à 10 %. Enfin, l'article 4 diminue les taux de retenue à la source en matière de redevances, tout en opérant une différenciation des plafonds applicables en fonction des catégories de revenus. Le taux de retenue à la source passe donc de 18 %, toutes catégories de redevances confondues, à 3 % s'agissant des redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales, à 5 % pour les redevances versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et à 10 % dans tous les autres cas. Notre pays a également négocié une clarification du champ des revenus compris dans les redevances. L'article 6 exclut ainsi explicitement des redevances les rémunérations de services « normalisés », c'est-à-dire ceux qui ne font appel qu'au savoir-faire usuel de la profession du prestataire. Cette stipulation est loin d'être anodine, en tant qu'elle acte la renonciation de l'Argentine à taxer les services rendus par une entreprise sans recours à un établissement stable sur le territoire argentin. J'en viens enfin aux stipulations relatives aux gains en capital. À la demande de la France, l'article 5 plafonne l'imposition dans l'État source sur les gains réalisés lors de la cession du capital d'une société lorsque le cédant détient une participation supérieure à 25 %, le taux maximum de retenue à la source est fixé à 10 %, tandis qu'il s'élève à 15 % dans les autres cas.

Certes, la diminution des taux de retenue à la source n'aura pas d'impact sur la charge fiscale totale des entreprises, puisque le cumul du prélèvement à la source argentin et du reliquat d'impôt français a vocation à égaler le montant de l'impôt que le contribuable aurait payé en France. Si le résultat de l'entreprise est déficitaire, en revanche, seul le prélèvement argentin subsiste. La diminution des plafonds de retenue aura alors un impact direct sur le niveau d'imposition des entreprises. L'insertion de plusieurs clauses du modèle France au sein de la convention franco-argentine a aussi été décidée. Sans entrer dans le détail de chaque dispositif, je tiens tout de même à souligner que ces différentes stipulations sécurisent le cadre juridique applicable aux relations fiscales franco-argentines, garantissent l'application du droit interne français et rendent conforme la convention de 1979 au modèle de convention de l'OCDE. Je relève également que la France a négocié la mise en place d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les volontaires internationaux, qui devrait concerner une quarantaine de personnes annuellement. Le troisième type de concession obtenue par la France concerne l'insertion au sein du protocole de la convention d'une clause de la nation la plus favorisée, dont la portée est relativement large. Notre pays disposait déjà d'une telle clause, mais celle-ci se limitait au régime des paiements effectués pour les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique.

indépendantes. Cette clause a donc une portée nettement plus vaste que la précédente. À cet égard, permettez-moi de vous signaler que, si la France avait bénéficié d'une telle clause dès 1979, nous n'aurions pas eu à négocier cet avenant, puisque les taux de retenue à la source pratiqués par l'Argentine auraient été revus progressivement à la baisse. Il me semble intéressant de préciser également que l'Argentine a conclu ce type de clauses avec de nombreux pays, ce qui a pu limiter nos marges de négociation. En effet, toute concession à l'égard de la France aurait dû automatiquement être accordée à d'autres partenaires. après vous avoir présenté les principales avancées obtenues par la France, il me faut maintenant vous exposer leur contrepartie, à savoir l'insertion d'une clause portant reconnaissance d'un établissement stable de services. L'Argentine souhaitait initialement taxer l'ensemble des services rendus par les entreprises françaises sur son territoire, sur une base brute et sans condition de durée, par le biais de l'article sur les redevances. Dans la mesure où cette clause aurait été particulièrement préjudiciable aux entreprises françaises, les négociateurs français ont refusé de l'insérer Les négociations ont finalement abouti à la reconnaissance de l'établissement stable de services en l'absence de toute installation matérielle. En principe, le siège français d'une entreprise qui ne possède pas de filiales en Argentine dispose du droit exclusif de taxer les bénéfices, sauf si un établissement stable est caractérisé sur place. Il peut s'agir d'un établissement stable traditionnel, c'est-à-dire d'un bureau ou d'un atelier. Cependant, la clause négociée dans l'avenant reconnaît également l'existence d'un établissement stable en l'absence de toute installation matérielle en Argentine, dès lors qu'une entreprise rend des services pour une période cumulée représentant plus de 183 jours au cours d'une année. Si un tel établissement stable est constitué, l'Argentine disposera du droit exclusif de taxer les bénéfices qui s'y rattachent. Cela étant, l'impact fiscal de cette disposition devrait rester limité, puisqu'elle ne concernerait qu'une trentaine d'entreprises sur les 250 qui exercent une partie de leur activité en Argentine. en Argentine. Les prestataires français qui interviennent plus de 183 jours par an sur un territoire finissent de toute façon par y constituer une installation fixe, donc un établissement stable ... Enfin, d'un point de vue budgétaire, je n'ai malheureusement pas pu obtenir de données chiffrées sur la perte de recettes fiscales pour le Trésor public. L'administration fiscale m'a toutefois indiqué que ces dernières devraient rester très limitées. Pour conclure, le nouvel équilibre conventionnel résultant de la signature de cet avenant est globalement avantageux pour notre pays. tenu de l'asymétrie de nos échanges économiques avec l'Argentine, la réduction des taux de retenue à la source sera très bénéfique au Trésor public, tout en améliorant la position concurrentielle de nos entreprises sur le territoire argentin. En parallèle, la reconnaissance d'un établissement stable de services ne devrait pas entraîner de préjudice fiscal de grande ampleur. Enfin, il convient de saluer la clarification opérée dans un certain nombre de cas, conduisant à sécuriser l'application de dispositifs de droit interne.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui entend élargir et actualiser dans le domaine fiscal les accords qui prévalent entre la France et l'Argentine depuis la convention du 4 avril 1979, modifiés par un avenant en date du 15 août 2001. Plus globalement, l'Argentine, membre du G20 et candidate à l'OCDE, a toujours été un partenaire majeur de la France en Amérique latine. La France, quant à elle, a toujours été aux côtés de l'Argentine, en matière tant de développement social et culturel que de développement économique : elle est le dixième fournisseur de l'Argentine et le quatrième parmi les pays européens, derrière l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Aussi, même si nous nous interrogeons sur les raisons qui ont justifié d'attendre une année avant de signer le décret de présentation de l'avenant nous ne pouvons qu'accueillir favorablement ce projet de loi ; il s'inscrit dans la logique de nos histoires respectives et a pour vertu, et non des moindres, d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Plus précisément, cette convention fixe les règles de répartition du droit d'imposer entre la France et l'Argentine en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et tend à rationaliser les doublons d'imposition qu'induirait l'application des législations fiscales nationales sur les différentes catégories de revenus qu'elle vise. Même si certaines conventions tendant à éviter les doubles impositions, conclues ultérieurement par l'Argentine avec d'autres États partenaires, fixent pour ces mêmes revenus des plafonds de retenue à la source inférieurs à ceux que prévoit la présente convention, force est de constater que le nouvel équilibre conventionnel devrait se révéler globalement favorable aux intérêts économiques français, notamment par l'introduction de la nouvelle clause de la nation la plus favorisée. En permettant à la France de bénéficier de taux de retenue à la source les plus bas possible, cette disposition paraît bénéfique pour les activités françaises. À l'avenir, notre pays bénéficiera donc automatiquement du traitement plus favorable que l'Argentine serait susceptible d'accorder à un autre État en matière de revenus passifs- intérêts, dividendes et redevances -, de gains en capital, de revenus de professions indépendantes ou d'établissement stable. L'insertion de cette clause constitue une concession significative, garantissant que la France bénéficiera toujours des taux les plus favorables octroyés par l'Argentine à ses partenaires. Ce texte est enfin l'occasion de souligner deux points sur lesquels je souhaite appeler votre attention. la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2020 élargit la notion d'établissement stable à nombre de situations qui visent l'économie numérique, avec des potentialités d'application plus larges. Il s'agit là d'enjeux dont la France doit absolument se saisir,

Il serait fastidieux que je reprenne à mon tour l'inventaire de ces arguments. Je souhaite, à l'inverse, que nous prenions un peu de recul et que nous mettions ce texte en perspective, notamment au regard de la politique fiscale du Gouvernement. Gouvernement. Depuis 2017, la majorité présidentielle s'est engagée à lutter contre la fraude fiscale et à renforcer le socle d'impositions de la France sur son propre sol et à l'étranger.

C'est à tous ces niveaux que nous avons porté nos efforts pour lutter contre la fraude et faire en sorte que tous les impôts dus en France soient acquittés par les contribuables sur le territoire de la République. Reste que tous ces outils, si précieux soient-ils, ne trouvent leur justification qu'à travers cette brique fondamentale de notre modèle fiscal que sont les conventions fiscales bilatérales. Celles-ci doivent être négociées ou renégociées régulièrement pour suivre les évolutions de nos droits nationaux et pour éviter les doubles impositions qui risquent de se multiplier à mesure que notre droit fiscal se complexifie. L'avenant que nous examinons ce matin se place dans cette logique. Il permet de mettre à jour la convention fiscale qui lie la France et l'Argentine- pays qui nourrissent depuis des années un étroit partenariat économique - et de la rendre plus favorable à notre C'est pour obtenir une réduction des taux de prélèvement à la source appliqués en Argentine que la France a souhaité renégocier cette convention, entre les mois de mai et décembre 2019. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, cette convention a notamment permis trois avancées considérables pour la France l'insertion d'une nouvelle clause de la nation la plus favorisée, la réduction des taux de retenue à la source, l'insertion de clauses spécifiques pour que notre pays puisse continuer à optimiser l'application de sa propre législation fiscale dans un certain nombre de cas. nombre de cas. La clause de la nation la plus favorisée est un outil très efficace, grâce auquel la France bénéficiera automatiquement du traitement fiscal le plus favorable accordé par l'Argentine à l'un de ses partenaires, que ce soit pour les gains en capital ou les revenus passifs. Les taux de Les taux de retenue à la source pénalisaient les investissements des entreprises françaises et grevaient à long terme les recettes du Trésor public. La diminution de ces taux profitera largement à la France. Elle concernera les dividendes ou les gains en capital, en cas de participation substantielle dans une société, mais également les intérêts qui seront ramenés à un taux proche du modèle de convention de l'OCDE. Enfin, l'avenant réduira les taux de retenue à la source concernant les redevances, en fonction des biens ou des oeuvres concernés. En contrepartie, la France a concédé au Gouvernement argentin une clause reconnaissant l'existence d'un établissement stable pour les entreprises de services intervenant plus de 183 jours en Argentine. Là encore, cette contrepartie sera limitée en ce qu'elle ne concernera qu'une trentaine d'entreprises. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera ce texte, comme nous y invite le rapporteur. Il continuera de soutenir le chantier entrepris par le Gouvernement pour renégocier l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Avec la convention multilatérale signée avec l'OCDE, qui permet de fixer des règles générales d'imposition, ce texte clarifiera la situation fiscale applicable entre la France et l'Argentine et encouragera cet effort de simplification et d'harmonisation.

vin, boeuf, soja ... -et ses sportifs. C'est une grande nation, à la fois du football et du rugby, avec des performances de classe mondiale dans les deux sports, le tout sur un air de tango ! Cet avenant à la convention fiscale de 1979 devrait renforcer la position des entreprises françaises implantées à la réduction de la taxation des revenus du capital. L'imposition de certains dividendes passera ainsi d'un plafond de 15 % à 10 %, et celle des intérêts de 20 % à 12 %. Les exportateurs français devraient alors être mieux avantagés par rapport aux concurrents internationaux, bénéficiant de conventions plus favorables et, surtout, plus récentes. Les jeunes salariés en volontariat international en entreprise seront quant à eux exonérés d'impôt sur le revenu. On ne peut que regretter la faiblesse relative des relations commerciales entre nos deux pays. Comme le rappelle l'étude d'impact, la France n'est que le quatrième fournisseur européen de l'Argentine, derrière l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Réciproquement, l'Argentine est pour nous un partenaire commercial moins important en Amérique latine que le Brésil, le Mexique ou même le Chili et le Pérou. L'un des points importants de l'avenant consiste en l'introduction de la clause de la nation la plus favorisée, règle bien connue du commerce multilatéral, popularisée en son temps par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et emblématique du principe d'équité des échanges.

Pour terminer sur une note originale, permettez-moi d'évoquer le cas de la truffe argentine, surnommée là-bas le « nouvel or noir ». Sa production est en plein essor. Destinée en grande partie à l'exportation, elle fait l'objet d'une méthode de récolte chronométrée et de conservation sous semi-vide, afin d'être exportée vers l'Europe et l'Amérique du Nord, sans que ses qualités gustatives soient altérées. La truffe du Nouveau Monde entend tirer bénéfice d'une commercialisation en contre-saison. Peut-être cette production contribuera-t-elle à relancer les échanges commerciaux, alors que la pandémie touche durement l'Amérique latine comme l'Europe ... En conclusion, en dépit de sa portée relativement limitée, cet accord comporte des éléments de progrès par rapport à la situation actuelle : le groupe du RDSE est favorable à son approbation.

Ici, il n'y a nulle ambiguïté. Sur dix articles, le score est sans appel : neuf à un, la France semble l'emporter haut la main ! Excellent ! Bien qu'il n'y ait pas de contentieux entre les deux États, le gouvernement français a jugé bon de diminuer les ressources fiscales argentines pour en récupérer autant. Certes, les finances publiques françaises sont en difficulté, on le sait, mais une analyse de la situation économique et sociale du peuple argentin aurait peut-être dû nous inspirer plus d'égards.

Les premiers bénéficiaires de cet accord seront notamment les grands groupes français qui se trouveront en situation de concurrence significativement avantagée. À cet égard, l'article 7 de l'avenant prévoit que la France bénéficiera automatiquement du traitement le plus favorable que l'Argentine accorderait à autre État.

la taxation des établissements stables, mais uniquement de services, seulement sur les bénéfices nets, à partir de 183 jours : c'est aux antipodes de la volonté initiale de nos partenaires argentins ! Pourtant, cette affaire s'est réglée en un seul tour de négociation, et pour cause : les bailleurs privés et la troïka maintiennent une pression constante sur le pays depuis soixante ans. Pour quel résultat ? Pour la neuvième fois de son histoire, le 22 mai dernier, l'Argentine a encore fait partie des six pays à avoir renégocié sa dette ou à avoir fait défaut en 2020. conséquence, ses créanciers, dont BlackRock, ont refusé la première offre de restructuration de la dette proposée par le gouvernement argentin. Ils n'ont pas voulu d'une réduction de 5,4 % du principal et de 62 % des intérêts.

contracté par l'ancien gouvernement libéral de Mauricio Macri auprès de cette même institution. Ce dernier s'extasiait alors devant l'ex-patronne du FMI en ces termes : « Je dois avouer qu'avec Christine nous avons entamé une grande relation depuis quelques mois, nous espérons que cela marchera et qu'au final l'Argentine tout entière tombera amoureuse de Christine. » L'avenir nous le dira Je ne sais pas si un Argentin s'est épris de « Christine », mais nul doute que tel n'est pas le cas du nouveau chef du gouvernement, qui doit désormais soustraire son pays au joug du FMI. Comme d'habitude, l'institution a déclaré avoir pour objectif final d'« aider l'Argentine à renforcer sa croissance et sa stabilité, générer de l'emploi, réduire la pauvreté ». Cette renégociation doit pourtant s'accompagner d'un programme économique. Nul doute que sera une nouvelle fois imposée à l'Argentine une cure d'austérité sous la forme d'un programme d'économies structurelles, peu susceptible de faire redémarrer une économie prise dans une spirale inflationniste, combinée à une récession chronique. Nous nous abstiendrons donc sur cet accord, qui aurait dû, selon nous, prendre en compte la réalité économique et sociale de l'Argentine et reposer, surtout, sur des principes de solidarité.

et les gains en capital. Pour bien mesurer les enjeux de cet accord, il faut rappeler que la France a longtemps figuré parmi les premiers investisseurs en Argentine, avant que la crise de 2008 ne change la donne. Aujourd'hui, selon les données de la Banque de France, confirmées par celles de la Banque d'Argentine, l'Argentine est la quatrième bénéficiaire de nos investissements directs en Amérique latine, cependant loin derrière le premier, le Brésil. La France figure ainsi au huitième rang des investisseurs étrangers en Argentine et au quatrième rang des investisseurs européens, mais loin derrière l'Espagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse. Quant aux investissements argentins en France, ils restent faibles, cela a été dit. L'Argentine est le fournisseur de la France. Dans ce contexte de déséquilibre entre la présence des entreprises françaises en Argentine et une moindre présence argentine en France, l'abaissement des niveaux de fiscalité prévu dans l'avenant jouera en faveur des intérêts économiques français et améliorera la position concurrentielle de nos entreprises sur le territoire argentin.

de l'adapter au paysage actuel de l'économie mondialisée, et, d'autre part, d'intégration des pays émergents et en voie de développement au sein d'un système fiscal initialement élaboré sans leur participation. Le 19 avril 2018, nous adoptions le projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion des bases d'imposition et le transfert de bénéfices liés aux stratégies d'optimisation des grands groupes mondiaux tirant parti des différences entre les régimes fiscaux nationaux. Les pertes de recettes liées à ces optimisations fiscales sont estimées à un montant compris entre 100 milliards et 240 milliards de dollars par an, soit entre 4 % et 10 % des recettes de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à l'échelle mondiale. Si les dispositions de la convention multilatérale visaient principalement à s'assurer que les bénéfices étaient imposés là où s'exerçaient réellement les activités économiques qui les engendraient, en luttant notamment contre l'utilisation abusive des conventions fiscales et le contournement artificiel du statut d'établissement stable, tout en améliorant les modalités de règlement des différends entre États en cas de double imposition, ce texte nous avait conduits cependant à exprimer de nombreuses craintes, qui demeurent d'actualité trois ans plus En effet, nous déplorions que la question de la fiscalité du secteur de l'économie numérique ne fût à l'époque que peu abordée dans toutes les conventions. La raison est pourtant connue : les divergences entre les États sur la question de la taxation des géants du Net ont empêché

Cette absence de consensus montrait que la communauté internationale était loin, voire très loin de mettre en place un dispositif commun. Nos craintes étaient fondées, car, trois ans après, nous avons assisté à la fin des grandes ambitions d'un groupe de travail dénommé, coprésidé

de l'opposition des États-Unis et du blocage d'un certain nombre de pays européens. Pour avancer sur ce sujet, il faut que l'Union européenne soit maintenant plus ambitieuse et qu'elle propose une refonte de la notion d'établissement stable, adaptée à l'économie numérique, à l'instar des avancées récentes sur ce sujet de la part de juridictions internationales et, en décembre dernier, du Conseil d'État. Enfin, l'enjeu de la coopération internationale en matière de fiscalité est bien de régler est bien de régler la contradiction entre une économie qui facilite la mobilité des marchandises, des services et des capitaux et un ensemble de réglementations fiscales segmentées, sur des territoires délimités, permettant tous les évitements des prélèvements. Or on continue ici à voter des avenants aux conventions fiscales bilatérales à un rythme soutenu, sans que la situation change véritablement à l'échelle internationale, ce qui met en évidence

Ce texte, cela a été rappelé par notre excellent rapporteur Vincent Delahaye, vise notamment à soutenir les quelque 250 entreprises françaises présentes en Argentine. Avec un peu moins champions du monde, un petit effort n'est donc pas malvenu. Les entreprises de plusieurs autres pays européens présentes en Argentine ont actuellement des taux de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, les redevances et les gains en capital inférieurs aux taux prévus par la convention de 1979, que nous revisitons complètement. Il s'est donc agi pour la France de remettre ses entreprises sur un pied d'égalité- pour une fois

argentine. L'Argentine est perdante dans cette convention fiscale, cela a été dit, mais n'est-ce pas l'agriculture française, derrière, que l'on menace en autorisant l'approbation de tel ou tel accord, dont nous ne voulons pas ici ? Revenons-en à la fiscalité. Le taux de taxation des dividendes est réduit de 15 % à 10 %. Il est en revanche maintenu à 15 % si le bénéficiaire détient moins de 25 % de la société qui paie les dividendes pendant un an.

vont malgré tout dans le bon sens et vont permettre d'encourager les investissements français en Argentine, ce qui est une très bonne chose pour nos entreprises, pour le rétablissement de notre balance commerciale, mais aussi pour l'économie de ce pays, qui en a besoin.

Au premier semestre 2020, au début de la crise sanitaire, la pauvreté touchait plus de 40 % de la population argentine. À titre personnel, mais aussi en tant que membre du groupe d'amitié

l'Argentine est très certainement le plus européen des pays d'Amérique latine. Depuis de nombreuses années, la France entretient d'excellentes relations avec ce grand pays, que ce soit sur le plan diplomatique, culturel ou économique. Qui dit relations économiques dit échanges de biens et de services et autant d'aventures entrepreneuriales de part et d'autre de l'Atlantique. Les questions fiscales posées par ces échanges relèvent d'une convention signée en 1979. Cette convention, déjà amendée en 2001,

la réduction des taux de retenue à la source ; l'insertion de clauses du modèle France ; la conclusion d'une clause de la nation la plus favorisée. Je ne m'attarderai pas sur les deux premières mesures, dont les aspects techniques ont déjà été rappelés par le rapporteur. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je me contenterai d'évoquer la clause de la nation la plus favorisée. Cette clause prévoit que la France pourra bénéficier, dans de nombreux domaines, des clauses plus avantageuses que l'Argentine concédera à d'autres pays que le nôtre, sur les revenus passifs ou les revenus des indépendants, par exemple. Il s'agit d'une avancée notable pour la France, qui ne bénéficiait pas, jusqu'à présent, de clauses aussi avantageuses que d'autres pays de l'OCDE, tels que l'Allemagne et l'Italie. Désormais, toute amélioration dans ces domaines profitera aussi aux 15 000 ressortissants français qui vivent en Argentine, ainsi qu'aux 250 entreprises françaises qui y exercent une part de leurs activités. C'est un choix courageux de la part de l'Argentine, dont la situation économique demeure très fragile. En effet, face au poison de l'inflation, l'Argentine doit sans cesse résister à ses penchants protectionnistes et isolationnistes. Cette volonté de renforcer les relations avec ses partenaires étrangers prouve qu'une nation peut aussi combattre ses démons par l'ouverture au monde. Elle va à l'encontre d'une vision moribonde et fermée de la souveraineté économique. Ce n'est pas rien pour un pays qui n'a jamais réussi à retrouver la place de premier plan qu'il occupait dans le commerce international il y a plus d'un siècle. C'est surtout beaucoup pour un pays qui a dû se déclarer en cessation de paiements en 2001 et qui est alors entré dans une crise économique terrible, dont il ne s'est pas encore relevé. Son endettement public s'élevait alors à 60 % de son PIB. Alors que nous devrons, dans les toutes prochaines années, mettre en oeuvre des politiques ambitieuses pour désendetter et pour réindustrialiser notre pays, le cas de l'Argentine peut nous donner matière à réflexion. En tout état de cause, nous nous réjouissons que nos pays renforcent leurs relations économiques.

de convention est à notre sens assez important, car il est logique de lutter contre les multiples impositions de l'ensemble des acteurs,

de travail et d'échanges qui sont de plus en plus pratiquées aujourd'hui par les acteurs économiques doivent conduire les responsables politiques à réadapter les modes de taxation.

en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (projet n°

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

(ACPR), qui seront principalement chargées d'accompagner ces professionnels, de fournir un service de médiation et de vérifier certaines conditions d'accès et d'exercice de leur activité. Lors de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 10 mars dernier, j'ai eu l'occasion de rappeler clairement ma conviction selon laquelle ce dispositif ne permettrait malheureusement pas de révolutionner la régulation de ce secteur,

D'autre part, ce dispositif ne mettra pas fin aux pratiques commerciales déloyales parfois observées dans ce secteur, compte tenu du fait que les associations professionnelles ne seront pas habilitées à exercer un pouvoir de contrôle sur leurs adhérents dans ces domaines. Ces deux limites ne sont pas dues à la volonté du législateur. Elles s'expliquent par les contraintes du droit de l'Union européenne. En dépit de ces deux regrets, cette proposition de loi constitue un premier pas, certes insuffisant, mais bienvenu. En effet, le dispositif est complémentaire des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui, compte tenu de la diversité et de l'atomicité du secteur, ne peut pas contrôler l'ensemble des acteurs, soit plusieurs dizaines de milliers d'intermédiaires. Le système proposé permettra de mieux accompagner ces intermédiaires, de vérifier que les conditions d'exercice sont remplies, ou encore d'offrir un service de médiation.

Premier apport : la possibilité pour toute association de notifier à l'ACPR et aux autres associations sa décision de refus d'adhésion.

Deuxième apport : la possibilité offerte aux associations de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d'intérêts,

Troisième apport : les dispositions visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d'assurance.

Nous avions privilégié ce mécanisme pour des raisons de fiabilité, l'Orias disposant d'un accès informatisé et donc sécurisé au casier judiciaire des dirigeants. Après un échange avec les acteurs concernés, il nous a semblé préférable d'écarter cette piste à l'heure actuelle. Celle-ci doit encore être approfondie par l'Orias pour être opérationnelle et gagnerait

S'agissant du démarchage téléphonique, le texte de compromis prévoit plusieurs ajustements par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture. Cette nouvelle mouture permet de rapprocher davantage le dispositif de l'avis du Comité consultatif du secteur financier financier publié en novembre 2019 sur le sujet. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas d'interdire le démarchage téléphonique des produits assurantiels, mais de créer un cadre législatif sécurisant pour le consommateur. Par conséquent, outre des modifications rédactionnelles, le texte prévoit des aménagements sur deux points. Premièrement, il introduit une distinction entre les appels sollicités et non sollicités. Ainsi, il est prévu que les dispositions encadrant le démarchage téléphonique, notamment l'obligation d'enregistrer les communications, ne s'appliquent pas

Monsieur le président,

que je suis avec intérêt depuis plusieurs mois, est le reflet de la volonté du législateur de mener à bien une réforme utile pour les courtiers comme pour les consommateurs. Au terme d'une lecture

à une proposition commune faisant l'objet d'un large consensus, ce que démontre son adoption par la commission mixte paritaire. Il m'importe de souligner clairement l'apport significatif

Entre les schémas d'escroquerie et le démarchage abusif, il existe un ensemble de pratiques très problématiques auxquelles il est nécessaire de mettre fin. Ce sera désormais possible. Cette nouvelle disposition, inspirée par les travaux du Comité consultatif du secteur financier, renforce l'information des assurés, interdit explicitement les « ventes en un temps » et précise les modalités de recueil du consentement du consommateur. Elle prévoit également une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années. Cela va permettre à l'ACPR et à la DGCCRF d'assainir le marché en détectant efficacement ceux qui, par leurs pratiques inacceptables, profitent et abusent de la fragilité de certains de nos compatriotes. Plus globalement, le Gouvernement salue la qualité du travail parlementaire, qui aura permis d'enrichir, de préciser et surtout d'améliorer ce texte. Je pense également aux dispositions ayant renforcé les garanties apportées aux courtiers dans leurs relations avec les associations professionnelles agréées, telles que la possibilité d'un retrait d'adhésion simplifié, l'obligation de motivation de tout refus d'adhésion ou encore l'ouverture d'un droit au recours en cas d'un tel refus. Je souligne en outre la pertinence des nouvelles dispositions renforçant les compétences des futures associations agréées, par exemple la possibilité qui leur est offerte de notifier à l'ACPR et aux autres associations une décision de refus d'adhésion. le Gouvernement approuve la décision prise par la commission mixte paritaire de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale concernant la vérification de l'honorabilité des salariés, dont je me souviens qu'elle a pu faire débat ici. Toutefois, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, le Gouvernement estime que l'Orias n'est pas en mesure d'assurer une telle mission, mais que les futures associations pourront utilement y contribuer en accompagnant les employeurs dans leurs démarches. D'autres apports de cette proposition de loi doivent être salués. Les futures associations professionnelles agréées permettront à la profession du courtage de s'organiser elle-même dans une logique de responsabilisation. Elles seront encadrées par des règles qui garantiront leur indépendance et leur impartialité. Elles fonctionneront en parfaite conformité avec le droit européen, car elles ne disposeront pas de mission de contrôle et ne constitueront pas des autorités compétentes au sens de la directive sur la distribution d'assurances. Elles auront des missions d'accompagnement. Les règles en matière de protection du consommateur sont pleinement mises en oeuvre. Elles permettront également de consolider notre réseau de courtage de proximité, qui compte beaucoup d'entrepreneurs individuels et de très petites entreprises qui contribuent à la vie de nos territoires. L'enjeu de cette réforme est de soutenir des professionnels qui peuvent parfois se sentir perdus quand il s'agit de se mettre en conformité avec une réglementation exigeante. Je pense par exemple à l'obligation légale de quinze heures de formation par an pour les courtiers d'assurance que nous impose le droit européen, ou encore à l'obligation de proposer un service de médiation pour le consommateur. Le périmètre de cette réforme, qui ne concerne que les courtiers et leurs mandataires, est un choix assumé de cette proposition de loi, que nous partageons. En effet, l'objectif n'est pas de surréglementer, mais d'agir uniquement lorsque cela est nécessaire. Ainsi, la proposition de loi vise spécifiquement les professionnels qui, à l'heure actuelle, ne bénéficient d'aucun soutien dans l'exercice de leur activité : les courtiers en assurance, les courtiers en opérations de banque et en service de paiement ainsi que leurs mandataires. L'ensemble des acteurs concernés par la réforme a jusqu'au 1 avril 2022, dans un an exactement, pour mettre en oeuvre ses dispositions dans les meilleures conditions possible et avec la plus grande sécurité juridique. Dans ces conditions, le Gouvernement apporte tout son soutien à cette proposition de loi, importante pour l'avenir de notre réseau de courtage ainsi que pour la protection des consommateurs français, et souhaite qu'elle puisse être promulguée dans les meilleurs délais. La parole

Le texte de compromis que nous nous apprêtons à voter définitivement ne constitue certes pas une révolution, le rapporteur l'a souligné. Cependant, il ouvre la voie à une amélioration de l'accompagnement des courtiers, ainsi qu'à un renforcement de la protection des consommateurs. À compter du 1 avril 2022, les courtiers d'assurances et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement auront l'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR. Ces associations joueront un rôle complémentaire de celui de l'ACPR et de l'Orias. Elles devront accompagner leurs membres, vérifier les conditions d'accès et d'exercice des activités et offrir un service de médiation, ce qui peut être fructueux pour les utilisateurs. Elles pourront par ailleurs refuser l'adhésion d'un courtier s'il ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession.

principalement par les nouvelles habitudes de consommation. En effet, dans un contexte de taux d'intérêt bas, nos concitoyens n'hésitent plus à faire jouer la concurrence pour réaliser des économies. Je me réjouis de l'élargissement des compétences des associations professionnelles, qui pourront non seulement notifier une décision de refus d'adhésion à l'ACPR, mais aussi formuler des recommandations à l'égard

été contraire au droit de l'Union européenne, qui n'autorise pas les associations professionnelles à contrôler leurs membres. Nous savons les dangers que cela peut comporter. Une autre avancée est l'amélioration de l'encadrement du démarchage téléphonique dans le domaine des assurances, avec le renforcement de l'information des souscripteurs ou adhérents éventuels, l'interdiction explicite des « ventes en un temps », ainsi que l'obligation de conservation des enregistrements des appels de vente. Pour ce qui concerne les courtiers étrangers qui interviennent sur le marché français au titre de la liberté de prestation de services ou de la liberté d'établissement- pas les Britanniques, bien sûr -, le droit de l'Union européenne nous impose de faire de l'adhésion à une association professionnelle une simple possibilité.

Pour autant, je suis convaincu que les courtiers étrangers seront nombreux à adhérer à une association professionnelle. Ils y auront tout intérêt, dans la mesure où ils y trouveront des renseignements, un encadrement, des gages de confiance. Je ne serais d'ailleurs

pour souligner à la fois l'ancienneté et la diversité des activités dites de courtage. À l'instar de mes collègues, je salue l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur la réforme du courtage en assurance et en opérations de banque.

a conservé plusieurs modifications adoptées au Sénat : la notification des décisions de refus d'adhésion, les recommandations en matière de bonnes pratiques commerciales et de prévention des conflits d'intérêts, mais aussi l'encadrement du démarchage téléphonique en produits d'assurance, qui reste l'occasion d'abus et de nuisances pour les consommateurs. Le courtage en assurance reste une activité peu réglementée et difficile à encadrer, car elle concerne des milliers d'acteurs, pas toujours domiciliés en France, face aux capacités de contrôle limitées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On peut attendre de l'adoption de cette proposition de loi que les secteurs du courtage en assurance et en opérations de banque s'organisent davantage, du fait de la nécessité d'effectuer des démarches supplémentaires d'agrément. Cela devrait renforcer la protection des consommateurs et le respect des règles de concurrence. L'obligation d'adhésion à des associations professionnelles agréées par l'ACPR permettra un meilleur contrôle, tout en conservant un système souple et la liberté d'établissement et de service. Son objectif, rappelons-le, est de mieux lutter contre certains abus, comme dans la vente de contrats d'assurance construction ou automobile, où des clients ont pu être abusés par des sociétés frauduleuses, parfois domiciliées à l'étranger. L'entrée en vigueur devrait avoir lieu d'ici un an, pour une réforme initialement proposée dans la loi Pacte en 2019. Le groupe RDSE votera donc en faveur des conclusions de la commission

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici réunis, après l'accord en commission mixte paritaire, pour traiter du sort des courtiers sans avoir l'assurance de la quelconque utilité des associations créées, ni même d'une quelconque capacité à protéger les consommateurs. Comme nous l'avions indiqué en première lecture, il ne s'agit pas d'installer des intermédiaires. Concurrentes entre elles, ces nouvelles associations ont un rôle flou et nous apparaissent sans réel objet. La proposition de loi cultive une ambiguïté sur les « recommandations » que pourraient formuler les associations agréées. Il a été reconnu à ce sujet lors de la réunion de la commission mixte paritaire qu'il « en résultera une généralisation des bonnes pratiques commerciales, même en l'absence de vérification ou d'audit organisé par l'association Pourtant, aujourd'hui, l'ACPR réalise des contrôles des bonnes pratiques commerciales. Elle a d'ailleurs mis en garde TCA Assurances pour ses pratiques commerciales « qui portent atteinte aux règles de bonnes pratiques de la profession ». En cause, le fait que ce courtier grossiste, spécialisé dans les structures subissant de plein fouet la crise sanitaire- restaurants, bars, discothèques ... -, a « anticipé [ ...] le renouvellement de contrats d'assurance souscrits auprès d'une société d'assurance opérant en France sous le régime de la libre prestation de services et dont il connaissait les graves difficultés financières ». Cette affaire nous inspire deux réflexions. Premier point : l'ACPR est une institution précieuse en matière de contrôle dont il aurait fallu renforcer les compétences et les moyens. Dans le même esprit, nous souhaitions accroître les prérogatives de l'Orias sur le contrôle de l'honorabilité. Cet amendement du Sénat a été écarté par la commission mixte paritaire au motif qu'il engendrerait un rallongement de la procédure d'embauche. La durée sera aussi longue si les associations agréées en ont la charge, et des risques sont présents s'il revient aux dirigeants d'attester sur l'honneur de l'honorabilité de leurs courtiers. prestation de services, ou LPS, dont nous avions fait grand cas lors de la première lecture, sont encore en cause dans cette affaire. Il faut le contrôle attentif de l'ACPR pour mettre au jour leurs dérives. La proposition de loi ne remédiera en rien aux errements de ces acteurs, qui s'évaporent parfois dans les paradis fiscaux, pour la simple raison que leur adhésion n'est pas obligatoire. Cette inégalité entre les acteurs français de l'assurance et les intermédiaires étrangers en LPS constitue à nos yeux un des motifs pouvant fonder une censure du Conseil constitutionnel. J'aimerais illustrer, à ce stade, grâce à un article de l'hebdomadaire, la détresse dans laquelle se trouvent les citoyens et les citoyennes tout comme les entreprises de construction de ce pays lorsqu'ils se rendent comptent des malversations de leurs assureurs. Nous sommes en 2016 à Drusenheim, dans le Bas-Rhin, où trois familles acquièrent, pour plus de 650 000 euros, un lot de trois maisons en vente en état futur d'achèvement. La livraison, prévue plus d'un an plus tard, est compromise deux mois après le début des travaux, lorsque le promoteur Building cesse de payer les maçons. Le chantier s'est arrêté, mais les familles ont continué de payer, car le promoteur avait réalisé de fausses attestations de fin d'étapes de travaux et autres certifications. Résultat, il a été placé en liquidation judiciaire. Les familles cherchent alors à récupérer leur garantie financière d'achèvement auprès de l'assureur choisi par le promoteur, obligé d'assumer le financement jusqu'à parfait achèvement des travaux.

L'histoire se répète. Les mêmes récits, les mêmes déceptions, souvent entre impuissance et abandon. Ce texte, à nos yeux, ne répond pas à ce fléau des intermédiaires étrangers en LPS qui gangrènent le marché français et laissent derrière eux des familles et des entreprises en proie au désespoir.

C'est le signe que nos deux assemblées sont capables, par-delà les clivages politiques, de se retrouver sur des positions communes lorsque l'intérêt général l'exige. Le texte final répond au double objectif affiché dans la proposition de loi initiale : protéger les consommateurs et clarifier le cadre réglementaire applicable aux courtiers. Réjouissons-nous que les améliorations apportées par la Haute Assemblée aient prospéré dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire. Ces améliorations sont significatives- même si elles sont insuffisantes, comme l'a souligné notre collègue Bocquet -concernant au moins trois points. Le premier d'entre eux réside dans le signal d'alerte envoyé au consommateur en cas d'infraction grave, par un intermédiaire, aux conditions d'adhésion à une association professionnelle. La possibilité pour toute association de notifier à l'ACPR ainsi qu'aux autres associations ses décisions de refus d'adhésion va incontestablement dans le bon sens. Nous nous en félicitons. Plus généralement, nous saluons la garantie apportée aux consommateurs grâce au surcroît d'information que leur offrent les systèmes d'adhésion à une association professionnelle et d'immatriculation auprès de l'Orias. deuxième avancée substantielle concerne la mission de recommandation donnée aux associations professionnelles en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d'intérêts. La formulation de ces recommandations devrait, dans les faits, favoriser une généralisation des bonnes pratiques commerciales. Dans le même sens, à savoir la protection du consommateur et de son intérêt, la validation par l'ACPR des statuts des associations devrait apporter une sécurité bienvenue. Enfin, s'agissant du démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d'assurance, la rédaction proposée par la commission mixte paritaire offrira une meilleure protection du consommateur, sans entraver les offres commerciales en cours. Nous pensons en particulier aux offres des comparateurs en ligne, qui sont les bienvenues en ce qu'elles offrent un choix plus large au consommateur. Il apparaissait ainsi utile de les sauvegarder. Le secteur du courtage étant soumis à un renouvellement très fréquent de ses milliers d'intermédiaires, le transfert à l'Orias du contrôle du casier judiciaire des salariés, que nous avions proposé en première lecture, n'a pas été conservé dans le Celui-ci restera donc aux mains des associations professionnelles. Nous en comprenons la raison au regard des échanges qu'ont eus les deux rapporteurs avec les acteurs concernés. Nous en appelons toutefois à la plus grande vigilance sur ce sujet, qui méritera une surveillance accrue compte tenu du nombre de faux documents susceptibles de circuler. Mes chers collègues, grâce à l'implication constructive de chacun des parlementaires et des deux rapporteurs en particulier, un premier pas est aujourd'hui réalisé. Certes, cela a été signalé à plusieurs reprises, des imperfections demeurent.

Vous connaissez les réserves que j'avais pu formuler devant vous il y a quelques semaines, au nom de mon groupe, réserves que je sais partagées par un certain nombre d'entre vous. Ce secteur d'activité gagnerait à être mieux encadré, mais l'option choisie, à savoir la création d'associations professionnelles à adhésion obligatoire, ne répond pas pleinement aux objectifs que cette proposition de loi s'était pourtant fixés, particulièrement en matière de protection des consommateurs. En effet, il convient de constater que la profession du courtage concerne un nombre très important d'acteurs, que les contrôles jusqu'alors exercés sont insuffisants et que les scandales récents ont mis en évidence la nécessité de mieux l'encadrer.

de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, chargée de vérifier la véracité des documents transmis à l'Orias et les pratiques des courtiers,

plutôt que déléguer purement et simplement ces missions à des associations agréées. En créant un intermédiaire supplémentaire entre professionnels et instances nationales de régulation, cette réforme semble manquer de cohérence à l'heure où l'on supprime en loi de finances des organismes de gestion agréés (OGA) jouant un rôle similaire sur un autre marché. Par ailleurs, ce texte, annoncé comme renforçant la protection des consommateurs, est loin d'apporter les solutions aux dysfonctionnements constatés, que ce soit en matière de libre prestation de services ou de pratiques commerciales déloyales. Cela a été souligné tout à l'heure par M. le rapporteur. De même, et j'avais déjà eu l'occasion de le souligner ici devant vous, cette autorégulation par des associations professionnelles favorisant de grosses entités de courtage

Je regrette une nouvelle fois l'absence d'étude d'impact qui aurait pu nous éclairer sur ce texte et nous indiquer en quoi un marché plus concentré pourrait profiter aux consommateurs. Je déplore également que le seul amendement sénatorial tendant à confier le contrôle de l'honorabilité des intermédiaires à l'Orias n'ait pas survécu à la commission mixte paritaire : malgré notre désaccord sur le fond, il me semblait important que ce point puisse être conservé dans la loi. ce texte consacre le recul du rôle de la puissance publique au lieu de lui donner les moyens d'exercer les missions et d'effectuer les contrôles nécessaires aussi bien pour les professionnels du courtage que pour la protection des consommateurs. Convaincu que d'autres options auraient pu être choisies pour encadrer ce secteur d'activité, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'abstiendra, comme en première lecture, sur ce texte.

d'une part, agir comme un tiers de confiance, afin de sécuriser une transaction, pour le client comme pour le fournisseur ; d'autre part, faire jouer la concurrence pour assurer une offre compétitive, tout en se rémunérant sur la bonne mise en relation de l'offre et de la demande. Son utilité doit donc être appréciée à l'aune de cette double valeur ajoutée. C'est aussi à cette aune que nous devons apprécier la pertinence du texte que nous examinons aujourd'hui. En effet, la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement manquera sa cible si elle ne permet pas de gagner sur les deux tableaux : la confiance, d'une part ; la compétitivité, d'autre part. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer en première lecture, je crois que le dispositif prévu par cette proposition de loi va dans le bon sens. Les associations professionnelles à adhésion obligatoire, agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, apporteront lisibilité et transparence aux consommateurs. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire, réunie le 10 mars dernier, soit parvenue à un accord sur le texte. Cet accord prouve le rôle constructif du Sénat dans la navette parlementaire, d'autant que plusieurs des amendements que nous avions votés ont été conservés dans le texte final. Surtout, il consacre l'aboutissement d'un travail de longue haleine, puisque les dispositions de cette proposition de loi avaient déjà été adoptées lors de l'examen du projet de loi Pacte voilà maintenant plus de deux ans.

de loi n'augmentera pas les prix. En effet, comme je l'ai déjà évoqué lors de la première lecture, la création des associations professionnelles à adhésion obligatoire entraînera mécaniquement des surcoûts pour les acteurs de la profession. Le risque existe que ces surcoûts soient ensuite répercutés sur le consommateur final. Mais il est également possible que la clarification des offres disponibles sur le marché renforce les acteurs les plus solides et leur permette donc d'améliorer leurs marges. Ces acteurs pourraient alors absorber les surcoûts en question sans avoir à les répercuter sur les consommateurs en augmentant leurs prix. Le texte atteindrait alors son double objectif. Malgré ce point de vigilance, le groupe Les Indépendants approuve largement le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. La parole est

des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d'intérêts. Même si cela reste dans la limite de ce que le droit européen autorise, cette amélioration permet de limiter en partie des contre-effets délétères induits par la réforme proposée. cette mesure ne nous semble que partielle au regard du fort risque de conflits d'intérêts qui demeure. La protection du consommateur ne nous semblait aucunement garantie. Le texte encadre désormais mieux le démarchage téléphonique en matière de distribution. De nombreux abus ont été pour certains produits assurantiels. Cela dit, le spectre reste relativement étroit et assez peu ambitieux en la matière, par rapport aux moyens que l'on aurait pu donner à l'Orias ou à l'ACPR pour l'exercice des contrôles nécessaires et une protection réelle des consommateurs. Si nous sommes conscients des perspectives d'amélioration, nous restons persuadés qu'il n'était nullement besoin de désarmer la puissance publique. Nous sommes également convaincus qu'il n'y avait aucune urgence à légiférer soudainement sur le courtage. C'est un sujet très complexe, dont il est difficile de maîtriser les tenants et les aboutissants. vous rappelle d'ailleurs que nous avons été privés d'une étude d'impact. Nous votons donc à l'aveugle une réforme dont il est impossible d'évaluer les effets ! Enfin, rappelons aussi que nous aurions largement préféré discuter de la place que prennent les assurances dans le soutien à la population au regard du contexte que nous connaissons tous.

Pour rappel, nous avions supprimé des centres de gestion lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Et voici que nous nous apprêtons à mettre en place une nouvelle obligation administrative pour les courtiers en assurances, obligation évidemment doublée d'une charge financière non productive

j'ai aussi pris conscience qu'il y avait un nombre considérable d'inscriptions et de résiliations d'inscriptions des intermédiaires en assurances et de leurs mandataires. aussi respecter des obligations de médiation, de formation et de garanties financières. Aujourd'hui, c'est peu suivi. Compte tenu de la taille moyenne des structures, ce n'est pas toujours facile. En revanche, j'espère voir cette proposition de loi protéger les assurés des courtiers étrangers

de loi que nous allons adopter prévoit donc que les courtiers en assurances dépendant de l'ACPR et immatriculés à l'Orias dès leur installation- l'adhésion est renouvelée chaque année -soient dorénavant adhérents à une association professionnelle à partir de 2022. Celle-ci assurera la médiation sur les litiges entre courtiers et clients, la formation des courtiers et l'information sur les nouvelles règles législatives ou normatives, ainsi que sur la garantie financière, moyennant une cotisation annuelle d'environ 500 euros. Le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques resteront à la charge de l'ACPR, et c'est tant mieux, et l'Orias continuera sans étendre ses compétences. Ces associations auront la possibilité de prévenir l'ACPR et les autres associations en cas d'irrégularités, mais elles pourront également formuler des recommandations encourageant aux bonnes pratiques et à la prévention des conflits. Étant donné cette dernière capacité qui leur est offerte, j'espère que de telles recommandations ne se transformeront pas en obligations, contraignant les professionnels du courtage de nouvelles normes franco-françaises dans les prochaines années. Car le risque est bien que la libre concurrence et la recherche d'innovations fassent les frais de ce formalisme normatif, comme on peut le voir dans beaucoup de domaines. Je le répète, j'ai été surpris du dépôt de dernière minute de l'amendement du Gouvernement tendant à imposer à tout intermédiaire, lors du démarchage des assurés, d'enregistrer la conversation téléphonique et de la conserver pendant deux ans.

du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.